et Social Européen. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, hier, le Président de la République s'est rendu à Mulhouse afin d'évoquer un sujet sensible, la lutte contre les communautarismes ou, selon la nouvelle sémantique, le « séparatisme religieux Cette prise de parole était attendue et elle est salutaire, car, oui, la menace que la radicalisation religieuse fait peser sur notre modèle républicain et laïc de vivre-ensemble est réelle.

Ce sont des réponses concrètes qu'il nous faut apporter aux situations quotidiennes qui se présentent aux communes, aux écoles, aux universités, aux associations, aux fédérations sportives ou encore aux hôpitaux ; la liste est encore longue Pour autant, monsieur le Premier ministre, j'ai eu, hier, la désagréable impression que le Président de la République s'engageait dans la voie de solutions passant, malgré passant, malgré les tentatives peu probantes de ses prédécesseurs, par un islam France. Or il y a un islam France, pratiqué par des milliers de musulmans, dans le respect des lois de notre République et de la laïcité. Cette dernière est là pour protéger les croyants comme les non-croyants contre les islamistes, islamistes, que la République ne doit donc pas institutionnaliser. Or, ce matin, le ministre de l'intérieur a précisé sur France Inter qu'il était prêt à accorder des moyens aux religions, loin des principes actuels de notre loi de 1905 ; cela nous paraît dangereux Aussi, monsieur le Premier ministre, quels sont véritablement les moyens que vous allouerez à la mise en oeuvre des annonces égrenées hier, afin d'apporter des réponses fortes aux menaces qui pèsent tant sur les Français de confession musulmane que sur notre unité nationale ? La parole

de sécurité. C'est la politique que nous menons dans le cadre de la reconquête républicaine, en particulier dans quinze quartiers. Nous en avons présenté le bilan d'activité- j'y reviendrai si nous en avons le temps démontre combien nous devons, tous ensemble, lutter contre l'organisation de ce séparatisme, c'est-à-dire contre les écosystèmes qui se créent et qui, au fond, cherchent à éviter, à esquiver la République. Le deuxième axe de ce plan, c'est la lutte contre les influences étrangères ; le Président de la République l'a abordé longuement hier. Le troisième axe consiste à redonner corps à la

ici, à commencer par moi, ne souhaite accorder des moyens, pour reprendre votre expression, au culte. Le principe même de la loi de 1905 doit être défendu et je le défends activement. Il n'est donc pas question de mettre en place des financements publics publics des cultes, quels qu'ils soient. Le principe de la laïcité est de faire en sorte que chacun puisse avoir le droit de croire, en en ayant les moyens ; nous devons contrôler cela. Le Président de la République s'exprimera de nouveau dans quelques jours, puis nous présenterons un plan d'action, sur lequel, j'en suis convaincu, nous nous retrouverons tous,

Des difficultés chez Renault, il y en a, certes, mais le groupe a cumulé 10 milliards d'euros de bénéfices au cours des quatre dernières années, et a versé le tiers de ceux-ci en dividendes aux actionnaires. Pour 2019, ce sont encore 312 millions d'euros de dividendes qui seront versés. On peut s'interroger sur la pertinence de ces choix.

et, surtout, pour engager autant qu'il est nécessaire la transition technologique et écologique indispensable. Or c'est désormais l'urgence absolue produire, comme le demandent les organisations syndicales, des véhicules multiénergies, hybrides ou électriques. En second lieu, la direction de Renault a fait des choix défavorables à la France,

l'État actionnaire a été défaillant ; en tout cas, il doit désormais veiller à ce que ce mouvement soit inversé et que des investissements de modernisation soient réalisés dans tous les sites français, que l'on regagne ainsi des capacités de production. Le préalable est de refuser la fermeture de sites pour engager leur mutation et la reconquête de l'emploi. Madame la secrétaire d'État, M. Le Maire a déclaré qu'il serait « vigilant

Ils sont emblématiques des défis que traverse aujourd'hui la filière automobile. Ces défis, je veux les rappeler parce qu'ils sont importants. Il y a trois défis structurels. Le premier, c'est la transition énergétique. Sachez-le, Renault a massivement investi dans cette direction, notamment en faveur du moteur électrique. Le deuxième, c'est celui du véhicule connecté,

défis imposent des investissements massifs ; c'est ce que vous constatez dans les comptes de Renault. Ces investissements consomment l'argent gagné et même au-delà, puisque l'on observe une trajectoire de cash négative. Le contexte conjoncturel ne facilite pas les choses : ralentissement aux États-Unis et en Europe, baisse en Chine. Or c'est dans ce contexte

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, il y a cinq jours, le parti La République En Marche a connu un politique anéantissant son dispositif électoral à Paris. Avec le Président de la République, vous avez alors désigné, en quarante-huit heures, la ministre des solidarités et de la santé comme candidate de substitution improvisée. Curieuse décision : en plein chaos de la réforme des retraites, de crise sans fin de l'hôpital public et de risque de pandémie du coronavirus, vous décidez de changer de ministre Votre gouvernement ne cesse de nous surprendre par sa légèreté, parfois par sa vulgarité, à l'instar de celle que votre ministre de l'intérieur a manifestée, ce matin, à l'égard de notre collègue Olivier Faure. Nous attendons, sur ce point,

Monsieur le Premier ministre, la France mérite que vous privilégiiez l'intérêt général plutôt que l'intérêt partisan ; nos concitoyens attendent donc votre réponse. La parole est à M. le Premier ministre.

... Je veux répondre à votre question de la façon la plus simple possible. J'ai effectivement dit, et je répéterai toujours, qu'Agnès Buzyn a été une remarquable ministre de la santé. Oh ! Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais j'ai le droit de vous donner mon avis !

combien Mme la ministre Agnès Buzyn a été, en la matière, engagée, compétente et remarquable. Elle a choisi de s'engager dans un combat politique.

souvent à l'extérieur, qui reprochaient à tel ou tel membre du Gouvernement une prétendue « déconnexion » par rapport au monde réel, puissent aujourd'hui s'étonner de ce qu'une ministre choisisse de défendre ses idées et son projet dans le cadre d'une élection municipale.

c'est un député compétent, qui a la triple caractéristique, qui ne me semble pas inutile en la matière, d'être médecin hospitalier,

Madame Cukierman, s'il vous plaît

l'action publique, dit ASAP, prévoit de libéraliser la vente en ligne de médicaments. L'objectif est d'encourager le développement de plateformes mutualisées et des locaux de stockage afin d'externaliser une partie des activités de vente des officines. Les médicaments ne sont pas des biens de consommation comme les autres ; 95 % de la profession et des Français sont opposés à une telle ouverture du marché. Le pharmacien est un professionnel de santé qualifié, disponible, à l'accès sans rendez-vous. Il est une porte d'entrée pour les soins primaires et la prise en charge des soins

de chiffre d'affaires. Or fragiliser le modèle économique des pharmacies pourrait conduire à des fermetures, notamment en milieu rural. En Allemagne et en Angleterre, un tiers des pharmacies sont menacées. Monsieur le ministre, la pharmacie est un maillon incontournable dans le circuit des médicaments, pour leur prise en charge sécurisée. Ce projet remettrait en cause le maillage territorial, avec une diminution du nombre de pharmaciens adjoints, estimée à 5 000. Avant la logique commerciale, nous devons préserver le lien de proximité. Cette réforme n'apparaît-elle pas contradictoire avec la volonté du Gouvernement d'améliorer l'offre de soins dans les territoires, notamment ruraux ?

un département qui, comme de nombreux autres, souffre déjà de la désertification médicale. Je comprends que c'est à ce titre que vous vous inquiétez de la possible disparition, demain, des pharmacies, qui sont des maillons essentiels de l'accès aux soins dans ces territoires sous-dotés. Votre question porte sur l'article 34 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, qui vise à simplifier, sans remettre en cause les équilibres de la vente en ligne, certains dispositifs de celle-ci. Je rappelle que la vente en ligne des médicaments est autorisée dans notre pays depuis quelques années, à la suite d'une décision européenne, et que les conditions d'application fixées par le projet de loi en limitent énormément la portée, parce que la France s'oppose à ce que de grandes plateformes, notamment étrangères, puissent, demain, vendre des médicaments aux Français dans des conditions de sécurité et de qualité qui ne seraient pas établies et qui viendraient mettre en difficulté le maillage

l'intention d'aller vers des plateformes de vente en ligne de médicaments comme Amazon- pour ne pas le nommer -ou d'autres. Le texte prévoit bien que cette activité restera sous la seule responsabilité du pharmacien d'officine, pour couper court à tout risque. J'espère que cette précision apaisera vos inquiétudes. Des amendements seront déposés pour clarifier les dispositions applicables et supprimer jusqu'à la notion même de plateforme. ces mesures de simplification ne doivent pas fragiliser les officines, dont la présence est indispensable sur le territoire. Je m'y engage, en cohérence, d'ailleurs, avec la politique de santé menée dans notre pays, depuis trois ans maintenant, par Agnès Buzyn, qui vise, au contraire, à donner de nouvelles missions aux pharmaciens d'officine sur notre territoire.

vous déclariez que « le site internet étant adossé à une pharmacie physique, les patients pourront si nécessaire se rendre dans une officine et échanger avec un pharmacien. Ceci constitue une garantie majeure

Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le nouveau président du Conseil français du culte musulman, M. Moussaoui, a rappelé, hier, que la majorité des musulmans de France veulent vivre leur spiritualité dans le strict respect des valeurs de la République. Il a ajouté que la volonté de faire reculer toutes les formes de communautarisme est en accord avec les idéaux de fraternité

Pouvons-nous déduire de la déclaration du Président de la République que votre gouvernement soutiendra notre proposition ?

d'être extrêmement mobilisés, aux côtés de l'ensemble des acteurs et des institutions publiques, pour faire reculer cet écosystème du séparatisme que nous connaissons. C'est ainsi que nous aurons fermé, en moins de deux ans, 15 lieux de culte, 12 établissements culturels et associatifs, 4 écoles, 150 débits de boissons, que nous avons mobilisé tous les moyens pour faire des contrôles et procédé à des redressements pour près de 19 millions d'euros dans ces quinze quartiers. Dès le mois de novembre dernier, j'ai demandé à l'ensemble des préfets que ce dispositif soit appliqué à l'ensemble du territoire national, parce qu'il a montré son efficacité et que nous devons bien évidemment agir.

Monsieur le ministre, vous avez soigneusement évité de répondre à la question que je vous ai posée. Elle n'était pourtant pas compliquée et était formulée clairement. Il faut donner un coup d'arrêt au communautarisme. La liberté religieuse n'autorise personne à exiger un traitement à part dans les hôpitaux, les écoles, les cantines, les services publics, les transports, les ateliers, les bureaux, les mairies, les piscines, les centres sportifs ni nulle part ailleurs. La Constitution est muette sur ce point. Il faut donc assumer de la compléter par une référence claire et connue de tous. Nous souhaitons le faire, non pas contre le Gouvernement, mais, si possible, avec lui. Le Sénat en délibérera à la fin du mois de mars prochain. Votre majorité devra ensuite prendre ses responsabilités pour permettre aux Français de se prononcer par référendum, après le vote, que j'espère positif, du Parlement. C'est ce que la Constitution prévoit, et c'est l'attente profonde de nos concitoyens.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances ainsi qu'à Mme la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Madame la secrétaire d'État, un an après l'échec de sa fusion avec l'allemand Siemens, Alstom vient d'annoncer son souhait de racheter Bombardier Transport, filiale ferroviaire du groupe canadien. Cette opération s'inscrit dans un contexte international de vive concurrence, en particulier avec le géant chinois CRRC, qui ne cesse de grignoter des parts de marché en Europe. Le rachat de Bombardier Transport par Alstom s'avère donc essentiel pour l'avenir de notre filière ferroviaire. Encore faut-il que la Commission européenne ne s'oppose pas à cette nouvelle initiative L'État français doit, bien sûr, soutenir sa filière ferroviaire au moment où la mobilité durable est devenue un enjeu majeur dans nos modes de déplacement. C'est pourquoi, madame la secrétaire d'État, nous serions heureux de connaître votre position sur ce projet de rachat et la stratégie de l'État pour accompagner cette opération. À ce sujet, que pouvez-vous nous dire des récents échanges du ministre Bruno Le Maire avec la commissaire européenne, Mme Vestager ? En outre, comme dans ma région des Hauts-de-France, des inquiétudes peuvent surgir chez les salariés de ces deux fleurons industriels, qui, finalement, exercent le même métier et pourraient craindre des compressions de postes ou des économies d'échelle, malgré un carnet de commandes bien rempli. Pour ma part, j'ai la conviction qu'ils sont le plus souvent complémentaires, comme sur les sites de production du Valenciennois, où Bombardier a 2 000 salariés et Alstom, 1 600. 600. Madame la secrétaire d'État, afin d'éclairer et de rassurer tous les salariés, comptez-vous demander à Alstom de communiquer rapidement sur son projet industriel et sur sa stratégie en matière d'emploi et, surtout, de tracer des perspectives pour tous nos sites de production en France ? La parole

Pourquoi ? Premièrement, au travers de ce rachat, Alstom va pouvoir renforcer son offre de produits, ses capacités de recherche et développement et ses capacités industrielles. Comme vous le dites très bien, celles-ci sont complémentaires.

sur le volet organisationnel, M. Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom, a indiqué très clairement que ce projet était un projet de croissance, qu'il reposait sur la complémentarité entre les sites- notamment, en France, de Bombardier et d'Alstom -et qu'il n'était pas question de le fonder sur la « recherche de synergies

La parole est à M. Frédéric Marchand, pour le groupe La République En Marche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la pédagogie étant l'art de la répétition, vous me permettrez, madame la secrétaire d'État, de revenir sur le dossier Alstom. Comme l'a dit ma collègue Valérie Létard, l'accord trouvé entre Alstom et la division transport de Bombardier pour le rachat de cette dernière doit permettre au groupe français de confirmer sa position de numéro 2 mondial de la construction ferroviaire. C'est bien évidemment une excellente nouvelle. Cette annonce prend bien évidemment une dimension toute particulière dans le département du Nord, et plus spécialement sur les deux sites voisins de l'arrondissement de Valenciennes celui d'Alstom, avec ses 1 355 salariés, à Petite-Forêt, et celui de Bombardier, à Crespin, qui compte 2 000 salariés. Tous deux ont leurs carnets de commandes remplis pour les quatre à cinq prochaines années, mais cette annonce pose irrémédiablement la question de l'avenir qui sera réservé aux deux sites. Alstom et Bombardier travaillent en consortium sur trois projets, dont le RER NG ou le M7, le train régional belge. La complémentarité géographique des deux groupes ainsi que celle de leurs produits sont des atouts mis en avant par le PDG d'Alstom pour « renforcer notre présence internationale ainsi que notre capacité à répondre à la demande toujours plus importante de solutions de mobilité durable ». Alstom et Bombardier, c'est aussi la participation à des projets innovants portés par le pôle de compétitivité de portée mondiale i-Trans, à Lille et Valenciennes, qui contribue à forger une identité exceptionnelle de ce bassin d'emploi en matière de transports.

Madame la secrétaire d'État, je vous sais, tout comme M. le ministre de l'économie et des finances, particulièrement attachée au développement de notre stratégie industrielle et de la dynamique de l'emploi. Aussi, quels éléments pouvez-vous nous apporter afin de garantir aux salariés que ce nouveau champion ferroviaire sera aussi le champion de l'emploi dans le département du Nord, qui a payé un lourd tribut à toutes les restructurations industrielles ?

S'appuyant sur des études scientifiques déjà disponibles, l'agence conclut, pour l'heure, à un manque important, voire à une absence de données scientifiques sur les effets biologiques et sanitaires potentiels de la 5G. Il apparaît, en effet, que deux inconnues principales doivent être levées. La première découle de l'absence d'études spécifiques relatives aux bandes de fréquences qui seront utilisées, notamment la bande La seconde tient à une des spécificités de la 5G, à savoir le ciblage du signal sur les utilisateurs, qui implique un temps d'exposition court, mais des niveaux d'exposition élevés. Des réponses à ces deux questions pourraient être apportées par le rapport final de l'Anses, prévu pour le premier trimestre 2021. Or la procédure d'attribution des fréquences aux opérateurs se déroulera très prochainement et les premiers déploiements devraient avoir lieu cet été. Il est pourtant évident que le bond technologique que constitue la 5G ne sera accepté qu'au prix d'une rationalisation du débat public, ce que ne permet pas le calendrier actuel. Madame la secrétaire d'État, pourrez-vous réellement tenir compte des conclusions du rapport de l'Anses, alors que les fréquences auront déjà été attribuées aux opérateurs et que la 5G aura commencé à être déployée ? Je rappelle, enfin, que les efforts de rationalisation doivent porter non seulement sur le volet sanitaire, mais aussi sur l'aspect environnemental. de l'énergie (Ademe), auditionné dans le cadre de la mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique, que j'ai l'honneur de présider, a ainsi déploré qu'aucune étude de l'impact environnemental du déploiement de la 5G n'ait été menée.

Parmi les dossiers abandonnés sur votre bureau par votre prédécesseur figure la question des pénuries de médicaments. « Elles se multiplient en France », titrait récemment un hebdomadaire. Un pharmacien résume ainsi la situation : « Les Les problèmes se multiplient, on ne sait même pas comment répondre aux patients qui veulent savoir pourquoi leur médicament n'est pas disponible, et on ne s'avance plus sur des dates de retour à la normale ! » À l'hôpital, l'indisponibilité de certaines classes thérapeutiques conduit à des pertes de chance inacceptables pour les patients. En raison du coronavirus, des inquiétudes se font jour sur l'approvisionnement en matières premières, excipients ou principes actifs, massivement importés depuis l'Asie. Je vous poserai donc une question en quatre points, monsieur le ministre. Pouvez-vous nous rassurer sur les résultats de l'analyse demandée à l'Agence nationale de sécurité du médicament afin d'identifier les risques possibles de ruptures d'approvisionnement liées au coronavirus ? Où en sommes-nous

Une expertise est-elle menée pour la mise en place d'un programme public de production de quelques médicaments exposés à des tensions d'approvisionnement ? Enfin, envisagez-vous de nouvelles initiatives, dans le cadre européen, pour remédier à une situation qui inquiète fortement nos concitoyens ? La parole

Cette démission intervient au moment où la crise du coronavirus fait son premier mort en France, où la réforme des retraites est quasiment dans l'impasse et où l'hôpital public traverse une crise profonde et durable. Je regrette en particulier que les mesures prises pour le personnel soignant concernent essentiellement les hôpitaux parisiens. Il y a de l'incompréhension et de l'étonnement, car être ministre du nouveau monde n'empêche visiblement pas de faire campagne pour les élections municipales : vous-même, monsieur le Premier ministre, faites campagne au Havre ; M. Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics, à Tourcoing M. Franck Riester, ministre de la culture, à Coulommiers ; Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, dans le quatorzième arrondissement M. Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, à Vernon ; Mme Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des armées, à Mont-de-Marsan ; et enfin, M. Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, à Marchenoir. Doit-on comprendre que, dans le nouveau monde, on peut être ministre à temps partiel et se présenter à une élection tout en annonçant à l'avance que l'on ne siégera pas comme maire ? Dans ce contexte, la démission de la ministre de la santé s'apparente encore plus à une désertion. Pour quelles raisons Mme Buzyn a-t-elle été obligée de démissionner du Gouvernement pour faire campagne à Paris ?

Madame la sénatrice, au nom de la majorité à laquelle j'appartiens, je vous remercie d'avoir cité les nombreuses villes dans lesquelles nous présentons des candidats de très grande qualité qui porteront nos couleurs à l'occasion des élections municipales.

en tant que ministre de la santé et des solidarités, je suis prêt à assurer la relève, à poursuivre l'action remarquable qu'elle a engagée dans le pays. Encore une fois, madame

Le 30 janvier dernier, l'Assemblée nationale examinait la proposition de loi de notre collègue député UDI, Agir et Indépendants, Guy Bricout, visant à allonger le congé de deuil après le décès d'un enfant. Le texte adopté était nettement en retrait des ambitions initiales de l'auteur, ce qui a suscité une émotion bien légitime

Techniquement, pour éviter les fourches caudines de l'article 40 de la Constitution, le Gouvernement doit s'engager sur un certain nombre de points.

porter à 25 ans la limite d'âge et à garantir le même droit pour les indépendants et les fonctionnaires ? Êtes-vous prêts à mettre en place une aide financière universelle pour les obsèques et de quel montant ? Êtes-vous favorables au maintien des prestations familiales, trois mois après le décès de l'enfant ? Ces points sont extrêmement importants et particulièrement attendus par les familles et les associations de soutien. soutien. Au-delà de ces aspects financiers, nous le savons tous, l'accompagnement social, administratif et médico-psychologique est tout aussi important pour les familles touchées par un tel drame.

Nous avons l'occasion, madame la sénatrice, avec vous, avec cette assemblée, avec la Nation tout entière, de bâtir un véritable accompagnement global pour ces familles à même de faire office de modèle en Europe.

périple de six mois à la rencontre des familles de France aux quatre coins du territoire. Le mot qui est le plus revenu lors de ces rencontres est celui de « solitude »

La parole est à M. Jean-Marc Boyer, pour le groupe Les Républicains.

Un rapport récent du Sénat vous propose de tenir compte de la réalité et de renouveler ce dispositif de soutien aux territoires ruraux. Les ZRR sont vécues comme un dispositif de justice, tout en respectant la libre administration territoriale. L'utilité du dispositif ne fait aucun doute, notamment en offrant une fiscalité adaptée aux acteurs économiques qui font le choix de la ruralité. Les exonérations fiscales, porteuses de leviers d'attractivité, soutiennent le tissu de proximité. votre politique, au service de métropoles, abandonne la proximité, pourtant essentielle en ruralité. Aussi la recentralisation étatique, voire étatiste, de vos décisions est-elle mal vécue par nos citoyens, dans nos villages. Ils y voient un pouvoir central qui gère d'en haut sans comprendre leurs besoins

de revoir une géographie prioritaire de la ruralité, comme l'a annoncé le Premier ministre lors du congrès des maires ruraux, en septembre dernier. Le travail des sénateurs

pour la réplique. Madame la ministre, nos villages de France, du plus petit au bourg-centre, font la richesse de notre pays.

une vague de témoignages d'athlètes abusés sexuellement dans leur jeunesse éclate au grand jour. Au-delà du patinage artistique, ce sont les mondes de l'escalade, du ski, du tennis et, maintenant, de l'équitation qui sont concernés, faisant des abus sexuels dans le sport un scandale qui renvoie irrémédiablement l'État à ses responsabilités. Parler d'« abus sexuels » me paraît à vrai dire bien pudique, puisqu'il s'agit plutôt, en réalité, de témoignages de pédocriminalité dans les clubs sportifs qui accueillent nos enfants dans nos territoires. Sachez, madame la ministre, que notre appui sera total tant il est urgent d'agir. J'aimerais à ce titre saluer l'organisation de la convention nationale sur la prévention des violences sexuelles dans le sport, qui se tiendra dans deux jours. Elle va dans le bon sens, puisque la pédocriminalité dépasse, hélas très largement le cadre du sport et que tous les acteurs sans exception doivent être mobilisés. De la même manière, la piste de l'élargissement du contrôle d'honorabilité aux bénévoles qui encadrent les mineurs dans le monde sportif paraît particulièrement opportune. Toutefois, le bénévolat n'est pas la seule faille du système. J'aimerais particulièrement attirer votre attention sur le modèle entraîneur-élève, qui structure largement le monde du sport et crée parfois une dépendance psychologique extrême, laquelle rend les mineurs vulnérables à la pédocriminalité, notamment lorsque l'entraîneur en vient presque à se substituer à la famille.

thématique et il est indispensable dans cette période de transparence salutaire que traverse le sport français. Comme vous l'avez dit, les témoignages des victimes, leur nombre, la gravité des faits, leur persistance dans le temps et l'impunité dans laquelle ils se sont déroulés sont aussi choquants que bouleversants. Ils le sont pour le grand public, pour le mouvement sportif, ainsi que pour l'État et ses agents. À ce titre, je tenais à remercier les agents de mon ministère de leur mobilisation en urgence pour écouter la parole qui se libère chaque jour. Après-demain, vous l'avez dit, Nicole Belloubet, Adrien Taquet, Marlène Schiappa et moi-même réunissons tous les acteurs, dont les parlementaires, pour une convention nationale sur la prévention des violences sexuelles dans le sport. Car la pédocriminalité, vous l'avez dit aussi, n'est pas un sujet spécifique au sport : en Europe, un enfant sur cinq en est victime. Le sport doit apporter sa pierre à l'édifice d'une société plus sûre pour nos enfants. Chacun doit s'approprier cette vigilance de chaque instant. Le pilotage des actions doit être mené main dans la main avec les collectivités et le mouvement sportif, afin de bâtir collectivement un plan national de prévention robuste et efficace,

Mais la vigilance devra aussi passer par des actions éducatives de formation et de prévention. Il s'agit de sensibiliser les enfants sur leur rapport à leur propre corps, chose qui n'est pas faite souvent dans notre société, y compris dans le cadre familial, et pour laquelle le sport peut jouer un grand rôle former les éducateurs sur les limites à poser et à tenir dans les relations entre les entraîneurs et les personnes entraînées que vous avez évoquées ; d'agir de manière constante pour dire qu'il est important de parler, de dénoncer et de signaler.

Monsieur le ministre des solidarités et de la santé, c'est avec une grande émotion que mon collègue Philippe Mouiller et moi-même vous posons cette question d'actualité, à la suite du drame qui s'est produit à l'hôpital psychiatrique de Thouars, dans le département des Deux-Sèvres, le jeudi 13 février dernier. Dans le cadre de son travail, Élodie, jeune infirmière de 31 ans, mère de deux enfants en bas âge, a succombé à un coup de couteau mortel donné par un patient. Ayons en ce moment une pensée pour sa famille, ses proches, ses collègues de travail et l'ensemble des salariés du centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, que le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie est venu rencontrer le lendemain du drame. Beaucoup de questions se posent quant aux conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Une enquête judiciaire est bien entendu en cours, mais nous pouvons d'ores et déjà pointer les nombreuses insuffisances qui touchent cet établissement. Comme partout en France, les services de psychiatrie sont engorgés, la sécurité n'y est plus assurée, la qualité des soins n'est satisfaisante ni pour les patients ni pour ceux qui les délivrent, les conditions de travail sont parfois indignes et le personnel est à bout de souffle. Ce drame met en lumière, monsieur le ministre, les insuffisances du nombre de personnels, le manque de moyens en matériels, ainsi que les besoins en termes de formations. Bien qu'élevées au rang de priorité par votre gouvernement dans le cadre du plan national Ma santé 2022, la psychiatrie et la santé mentale restent les parents pauvres du secteur de la santé, alors que le nombre de personnes prises en charge explose. Nous ne pouvons plus nous contenter de constats, de diagnostics, de conclusions, de rapports. Il convient maintenant d'agir de manière urgente et concrète. Monsieur le ministre, à la suite de votre prise de fonctions, vous avez prévu de vous rendre dans les prochains jours sur le site de Thouars. Le personnel du centre hospitalier appréciera votre démarche. Quelles sont les mesures d'urgence que vous pensez lui annoncer pour éviter que ce type de drames ne se reproduise ? La parole

mon histoire personnelle, il se trouve que, pendant mon internat de médecine à Grenoble, j'ai travaillé pendant six mois comme interne dans un service de psychiatrie. C'est émouvant ! J'y ai vu la difficulté de l'exercice au quotidien,

parfois des situations de dangerosité, dont les conséquences sont intolérables, je vous rejoins parfaitement sur ce point. Vous l'avez souligné, le délégué ministériel à la santé mentale s'est rendu sur les lieux. J'ai annoncé hier que je le ferai également, sans presse, pour rencontrer les équipes hospitalières, discuter et faire le point sur ce traumatisme, qui reste, je l'imagine, immense, quelques jours après le drame qui a touché cette jeune infirmière, mère de famille de 31 ans. Vous posez la question des moyens accordés à la santé mentale dans notre pays.

d'ici au début de l'été 2020. Des mesures importantes ont été prises et budgétées dans le cadre du dernier budget de la sécurité sociale. Je vous le garantis, le Gouvernement a pris à bras-le-corps le sujet de la santé mentale. J'espère que vous l'aurez compris, il s'agit aussi d'une question personnelle. La

les auditions des ministres. Ils ont abouti aux mêmes conclusions, vous nous en avez fait part, la psychiatrie reste le parent pauvre du secteur de la santé. La réalité est alarmante. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour revoir l'organisation de la santé mentale sur le terrain et donner les moyens budgétaires suffisants pour prendre en compte le quotidien de nos soignants. La

voilà que, dans un ciel passablement assombri, nous voyons arriver ce que j'appelle un « OSNI », un objet statistique non identifié. Il s'agit du revenu moyen par tête,

Dans ces conditions, comment les Français pourraient-ils vous faire confiance ? Ils ont bien compris que rien, absolument rien, dans ce projet n'est sécurisé. Nous considérons donc qu'il vous reste deux possibilités, monsieur le ministre : vous avez le choix entre une sagesse responsable qui vous amènerait à retirer ce dossier ou une obstination qui deviendrait coupable. Quelle voie choisirez-vous ? Madame la sénatrice Monique Lubin, vous avez parlé de confiance. Vous avez raison, c'est là tout l'enjeu. Dans le

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la mission d'information sur le thème : « Quel rôle, quelle place, quelles compétences des départements dans les régions fusionnées, aujourd'hui et demain ? »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 affaires économiques, la discussion de la proposition de loi visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace,

nous sommes appelés à voter, cet après-midi, un texte important : important, parce qu'il concerne un sujet stratégique pour l'avenir, la liberté du consommateur au sein de l'économie numérique ; important,

va au-delà de nos rangs, puisque c'est plus de la moitié des sénateurs qui l'a cosignée. Cela souligne une fois encore, s'il en était besoin, la spécificité de notre assemblée, où des majorités d'idées se dégagent par-delà les clivages politiques et où le mot « consensus » n'est ni un gros mot ni un vain mot. Ainsi, des parlementaires de tous bords se sont unis pour agir sur l'un des enjeux essentiels de notre temps, un sujet qui concerne la quasi-totalité de nos concitoyens, au quotidien, du soir au matin, sans même, souvent, qu'ils s'en aperçoivent, à savoir l'enfermement des consommateurs, sur internet, par quelques acteurs dominants, efficaces, puissants pourrait-on dire, trop puissants. Si le Sénat adopte ce texte aujourd'hui, il pourra s'enorgueillir d'avoir contribué à mettre ce sujet au coeur de la scène politique française et européenne. adresser mes remerciements appuyés et affirmer ma gratitude à tous mes collègues qui ont bien voulu s'associer à cette démarche inédite. En dépit de la qualité de leurs services et de leur contribution à l'innovation,

économique excessive de quelques-uns et la restriction de la liberté des consommateurs qui en résulte, ceux-ci ne pouvant plus faire jouer la concurrence par la qualité. Ne négligeons pas l'enjeu en question. Ce qui a fait l'efficacité du marché, c'est la concurrence la concurrence comme facteur essentiel de diversité de l'offre, d'accroissement de la productivité et d'intensité de l'innovation. Or ceux qui étaient hier des start-up sont aujourd'hui d'énormes entités économiques, qui abusent de leurs positions dominantes sur un marché où la taille est devenue essentielle. Et la tendance ne risque pas de s'inverser ! Malgré les scandales et les amendes à répétition- plus de 8 milliards d'euros d'amendes infligés à Google en Europe en trois ans -, les marchés financiers continuent d'accorder leur confiance à ces géants,

le commerce en ligne prend une place croissante dans les habitudes de consommation. Internet promettait d'être l'eldorado de la liberté : liberté d'entreprendre pour les entreprises, liberté de choix pour les consommateurs. Grâce aux smartphones, auxquels nous recourons de plus en plus pour accéder à internet, il est possible de consommer en tout lieu, à toute heure. Or, aujourd'hui plus que jamais, les smartphones sont régis par un duopole d'écosystèmes en silos : nous sommes dans les mains d'un duopole qui a toute latitude pour organiser comme il le souhaite la façon dont nous agissons en ligne. C'est comme si une entreprise mettait à fabriquer des postes de télévision qui ne nous laisseraient le choix que de regarder une seule chaîne ! Il n'est pas question de nier les bienfaits de l'économie numérique, qui est avant tout une fantastique opportunité pour nos entreprises, et un lieu bouillonnant d'innovations. Il n'est pas non plus question de nier la qualité des services apportés par les géants du Net, qui investissent beaucoup. Simplement, ils ont acquis un poids trop important, et, si nous n'agissons pas, tous les marchés numériques pourraient bientôt être constitués d'un duopole formé d'un géant américain et d'un géant chinois. Plus nous attendons, plus le choix des consommateurs est limité, plus l'innovation est corsetée, et moins nos entreprises se développent. Tant que nous n'agissons pas, les acteurs économiques- c'est logique et rationnel -n'ont aucune incitation à modifier leurs comportements. Tant que nous n'agissons pas, ils ont toutes les raisons de tuer la concurrence et d'enfermer le consommateur dans leurs écosystèmes Tant que nous n'agissons pas, c'est un signal de laisser-faire que nous envoyons, alors que la nécessité d'agir est chaque jour démontrée- et les rapports qui documentent page après page les effets induits par cette situation oligopolistique devraient nous y inciter ! Nous devons rééquilibrer les relations entre les grands d'internet et les utilisateurs

pourquoi ne pas attendre d'agir à l'échelle mondiale ? Et puisque Jeff Bezos et Elon Musk entendent rendre possible la vie dans l'espace, pourquoi ne pas attendre d'agir au niveau intergalactique ? Si je me permets ce petit détour par l'absurde,

cas à brève échéance ! Je crois profondément à l'Europe, mais le temps est à l'urgence. Souvenez-vous de la fameuse taxe Gafam ! Pendant combien de temps les gouvernements successifs ont-ils répondu aux parlementaires qu'il fallait agir à l'échelon européen, si ce n'est international ? Combien de temps perdu pour finalement se résigner à opérer au niveau national et ainsi mettre fin à un élément essentiel de la concurrence déloyale des géants du numérique ? En fait, monsieur le secrétaire d'État, nous sommes d'accord avec vous : il faut agir à l'échelle européenne. Et nous soutiendrons toutes les initiatives que vous pourrez proposer en ce sens. Mais, en attendant, pourquoi ne pas intervenir à l'échelon national ? Pourquoi prendre le risque d'une emprise toujours plus grande de quelques entreprises sur les marchés numériques, alors que nous avons le pouvoir de limiter la casse- pardonnez-moi cette expression Pourquoi faire preuve de tant de pudeur quand l'Allemagne, elle, a déjà publié un avant-projet de loi musclant le droit de la concurrence pour l'adapter à l'ère numérique ? Nous ne devons pas céder à la résignation. Agissons à la racine du problème en adaptant la régulation économique à l'ère des géants du numérique. Confions à un régulateur le soin de fixer un cadre, et même un cap, au marché.

tous les États membres ne partagent pas les mêmes points de vue. Vous le savez comme nous : le calendrier européen nous amènera au mieux en 2022, au pire en 2024. Et vous le savez comme nous : la pression parlementaire que nous exerçons par le biais d'envoyer un signal aux institutions bruxelloises. Ces dernières sont attendues sur ce sujet ; il faut qu'elles le comprennent ! Nous mesurons pleinement la difficulté de la tâche. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui à la Haute Assemblée d'adopter ce texte. Monsieur le secrétaire d'État, si le Sénat vote ce texte, la balle sera dans votre camp, et dans celle de nos collègues députés, pour inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ! Et, dans tous les cas, nous aurons l'occasion de rediscuter de ce sujet lors de qui contient des dispositions relatives au numérique, au droit de la concurrence et aux communications électroniques. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme l'a dit la présidente de la commission et première signataire de cette proposition de loi, nous examinons aujourd'hui un texte qui nous rassemble largement. Le groupe socialiste et républicain a tenu à y apporter d'emblée une contribution active, la fonction de corapporteur que j'ai le plaisir d'exercer. Ces travaux sont pour moi le prolongement de ceux que j'ai effectués dans le cadre de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, que j'ai eu l'honneur de présider et dont Gérard Longuet a été

La commission d'enquête avait souligné le manque de coordination et de visibilité de la stratégie gouvernementale en matière numérique. Nous avions relevé le fonctionnement en silos des ministères et l'absence de stratégie globale. Nous avions donc recommandé la création d'un forum temporaire pour remettre à plat la stratégie française en matière de souveraineté numérique, et l'élaboration d'une loi d'orientation et de suivi de la souveraineté numérique. Monsieur le secrétaire d'État, je me permets d'insister de nouveau sur ce point ; plus le temps passe, en effet, et plus je suis convaincu de la nécessité d'une telle démarche. Continuer à subir, procrastiner en invoquant moult raisons, c'est nous condamner à la « silicolonisation » de la France et de l'Europe, pour reprendre le néologisme parlant du philosophe Éric Sadin. J'en viens à la proposition de loi. L'enjeu qu'elle a pour vocation de traiter est celui du rééquilibrage de la relation entre les géants du Net, ou plateformes structurantes, d'une part, et les consommateurs, d'autre part. Elle prévoit, dans ses deux premiers chapitres, de confier à un régulateur la mission d'orienter le marché de telle sorte que des comportements dommageables ne puissent voir le promeut une logique de régulation,, et d'accompagnement des acteurs. La sanction n'est là que pour crédibiliser la régulation, mais l'idée est de ne pas avoir à y recourir. La célérité avec laquelle des comportements dommageables pour les concurrents et pour les consommateurs peuvent apparaître dans l'économie numérique justifie de compléter la régulation, celle celle du droit de la concurrence ou des pratiques restrictives de concurrence. La réglementation,, n'est en effet pas suffisamment réactive. C'est pourquoi il faut repenser la logique de l'action publique. C'est ce qui est envisagé dans la proposition de loi, avec deux points d'entrée que sont la neutralité des terminaux et l'interopérabilité des plateformes.

Mais le coeur de la proposition de loi est bien d'inventer de nouvelles formes de régulation des plateformes structurantes : une régulation plus agile, plus efficace, qui ne bride ni n'empêche l'innovation et qui permette de mettre un terme à la dynamique d'enfermement du consommateur que l'on constate aujourd'hui- Nous avons suivi l'avis du Conseil d'État, et les amendements adoptés en commission visent notamment à assurer la conformité de notre dispositif au droit de l'Union européenne. Sur ce point, la directive dite e-commerce, adoptée au début des années 2000, a montré son inadaptation au contexte économique nouveau. Cette directive consistait, entre autres, à limiter strictement la possibilité pour les États d'édicter des réglementations pesant sur les services de la société de l'information, afin d'en favoriser l'essor.

Vous le reconnaissez vous-même, il y a urgence à agir, et le Parlement dans son ensemble doit prendre ses responsabilités. Si, comme je le crois, la chambre haute adopte ce texte aussi largement qu'il a été cosigné, il ne tiendra qu'à vous et au gouvernement dont vous êtes membre de le faire voter par l'Assemblée nationale. De la sorte, la France aura donné l'exemple, comme l'Allemagne, d'ailleurs, dans un contexte européen où l'on sait que les calendriers de l'action publique effective sont toujours très longs et parfois préjudiciables, comme c'est le cas en l'espèce, aux économies nationales ! La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est à tous les utilisateurs de smartphones que nous nous adressons à travers la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Avec les smartphones, chacun est libre de communiquer, d'échanger et de consommer, où il veut, quand il veut. Comme le dit la publicité : le monde est à portée de main. Mais la réalité est que le monde est orchestré par deux acteurs, Apple et Google. Il est souvent difficile de s'en rendre compte, mais ces deux acteurs dominants possèdent toute la chaîne de valeur, des systèmes d'exploitation aux applications en passant par les magasins d'applications et, s'agissant d'Apple, la fabrication du terminal lui-même. Ils sont ainsi en mesure de verrouiller l'accès des entreprises à leur écosystème et d'y enfermer les consommateurs. Impossibilité de désinstaller certaines applications, impossibilité d'en installer certaines traitement discriminatoire des applications tierces par rapport aux applications « maison », sont autant de manières de brider la concurrence et de limiter la liberté du consommateur. Si le texte que nous examinons aujourd'hui était adopté, demain, ces comportements seraient sous le contrôle d'un régulateur dédié.

C'est ce que nous suggérons aujourd'hui de faire en passant du constat à l'action. C'est aussi à tous les utilisateurs de réseaux sociaux que s'adresse cette proposition de loi. Bien des échanges ont déjà eu lieu sur ce sujet dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus Nous pensons que l'interopérabilité des réseaux sociaux, comme celle d'autres plateformes, est un outil essentiel pour rendre le pouvoir au consommateur, lui permettre d'arbitrer entre diverses plateformes et de communiquer avec les utilisateurs d'autres plateformes. La proposition de loi rendrait possible, sous le contrôle de l'Arcep, l'émergence d'agrégateurs de comptes de réseaux sociaux, comme il existe aujourd'hui des agrégateurs de mails.

interdit le recours à des interfaces trompeuses, ces modes de conception des interfaces numériques qui orientent techniquement les choix du consommateur et le piègent de façon discutable. Généralement appelées, ce sont par exemple des cases pré-cochées relatives au paiement d'une assurance que l'on ne souhaite pas, ou le fait d'avoir toutes les difficultés du monde à se désinscrire ou se déconnecter d'un service. La proposition de loi tend également à renforcer le droit de la concurrence. Les seuils de déclenchement du contrôle des concentrations comprennent aujourd'hui de nombreux angles morts. dans le monde numérique, les géants américains et chinois, qui disposent d'énormes trésoreries, adoptent des stratégies d'acquisition à tout-va et passent entre les mailles du filet, ce qui éveille des soupçons légitimes sur ces acquisitions. Est-ce un phénomène dont les autorités de la concurrence doivent se désintéresser ? Nous ne le croyons pas, et nous proposons de rendre la vue à l'Autorité de la concurrence sur ces opérations, ne serait-ce que pour éteindre les soupçons ! Si une opération de rachat d'une entreprise active en France par un géant numérique devait poser un problème de concurrence sur le marché français, nous serions alors armés pour y répondre. En commission, nous avons tenté de déterminer un faisceau d'indices auquel l'Autorité de la concurrence pourrait avoir recours pour caractériser les géants du numérique. Car l'objectif est bien de viser les entreprises du numérique les plus importantes dans le monde et en Europe. C'est d'ailleurs un objectif qui irrigue l'ensemble de la proposition de loi : ne rajouter une « couche » de réglementation que là où c'est nécessaire et, ainsi, éviter d'imposer les mêmes règles à tous, des règles qui dans les faits ne peuvent être absorbées je veux souligner de nouveau le fait que nos partenaires allemands ont publié un projet de réforme du droit de la concurrence en vue de l'adapter à l'ère numérique. Monsieur le secrétaire d'État, cela me paraît un véritable encouragement à faire du couple franco-allemand le moteur de l'Europe sur ce sujet ! La parole

si nous devions en cet instant faire un bilan du développement de l'internet, nous y verrions deux mouvements paradoxaux : une promesse d'universalité empreinte d'ouverture et de neutralité, et une concentration continue encouragée par l'évolution de nos usages. particulièrement contribué à cette concentration, et parmi ceux-là l'utilisation des terminaux. Nous consommons désormais de l'internet prioritairement par le biais de mobiles et non plus des ordinateurs classiques. En privilégiant ce mode d'accès, nous conditionnons notre entrée dans le monde numérique à l'utilisation d'environnements logiciels qui offrent non pas un choix, mais seulement l'illusion d'un choix. Lorsque nous utilisons notre téléphone, nous nous glissons dans les contraintes du système d'exploitation et de ses applications préinstallées dont certaines limitent sciemment certaines fonctionnalités, voire préemptent nos décisions. Sans doute cette évolution est-elle d'abord le fruit de notre penchant naturel pour la commodité : plus il est facile d'utiliser un service, plus celui-ci devient puissant, de telle sorte que la commodité se révèle être un terreau propice au développement de positions dominantes. Cette mise en balance du confort procuré et de la liberté abandonnée ne saurait toutefois justifier, dans l'économie numérique, la mainmise croissante des systèmes d'exploitation sur l'accès aux contenus et aux services de l'internet. Cette situation, nous la constatons chaque jour. Elle ne fait qu'asseoir plus encore la domination des grandes entreprises du numérique, qui disposent d'une puissance de marché forte et persistante, de capacités de contrôle de l'accès et du fonctionnement du marché, d'économies d'échelle et d'effets de réseau très importants.

parfois soumises à des conditions contractuelles, avec des plateformes structurantes qui leur sont particulièrement défavorables et interrogent sur le partage de la valeur. Il y va de la valeur. Il y va enfin de notre souveraineté française et européenne. Je me réjouis de partager avec vous cette conviction commune. Je remercie le Sénat, et tout particulièrement Mme Sophie Primas, des travaux menés en préparation de l'examen de ce texte. Les thèmes abordés couvrent au fond trois enjeux stratégiques : la neutralité des terminaux, l'interopérabilité des plateformes et le contrôle plus efficace des concentrations. Ces enjeux décisifs sont au coeur de la réflexion du Gouvernement. Je veux d'abord rappeler que nous ne sommes pas dépourvus de leviers d'action à l'échelon national sur ces questions, que ce soit au travers du droit de la concurrence ou par le biais d'autres outils. Ainsi, le droit de la concurrence permet d'ores et déjà d'agir en matière de ventes liées. Il faut rappeler que la Commission européenne vient de condamner Google à une amende de plus de 4 milliards d'euros pour des pratiques de ventes liées de l'application Google Search et du navigateur de recherche Google Chrome, avec des pré-installations systématiques sur les appareils Android et Windows Mobile. Nous disposons en outre, le code de commerce, d'instruments en matière de pratiques restrictives de concurrence qui permettent par exemple à la DGCCRF de sanctionner des conditions commerciales manifestement abusives, les clauses créant un déséquilibre significatif au détriment d'une partie, les ruptures brutales de relations, et l'obtention d'avantages manifestement indus ou disproportionnés. C'est dans ce cadre que le ministre de l'économie a assigné Apple et Google devant le tribunal de commerce de Paris en 2017 et 2018 pour avoir soumis les développeurs d'application présents sur l'App Store ou Google Play à des obligations créant un « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties Des outils existent donc pour agir sur les questions légitimes soulevées dans le cadre de cette proposition de loi, et il convient que nous continuions de les mobiliser au maximum. Mais frapper juste, c'est frapper au bon moment, et bien souvent la régulation, c'est-à-dire celle qui constate et condamne les pratiques, est trop tardive et ne permet pas de corriger des situations de domination durablement ancrées. Comme vous le proposez, mesdames, messieurs les sénateurs, il faut que les régulateurs puissent orienter la manière dont sont conçus les produits et les services des plateformes structurantes, afin d'éviter qu'elles n'imposent une forclusion du marché. Toutefois, une régulation opérante n'aura de sens qu'à un niveau permettant d'appréhender efficacement les difficultés technologiques et juridiques que posent la taille et la complexité des géants mondiaux du numérique. Cet échelon, j'en suis persuadé, est celui de l'Union européenne. Quel État membre ou quelle partie de monde peut se targuer d'avoir infligé un total record de 8,2 milliards d'euros d'amendes en deux ans à Google pour abus de position dominante ?

À problème structurant, réponses structurantes : il est nécessaire de déployer une supervision et une régulation spécifiques pour les acteurs systémiques ayant une empreinte sur notre économie et notre démocratie. Cela

ainsi que de solides garanties juridiques, ce système devant s'appliquer à des acteurs dont la grande majorité sont établis hors de France. Je pense notamment aux règles harmonisées encadrant la mise sur le marché des terminaux, l'e-commerce, ou encore la prestation des services de médias audiovisuels. Pour l'ensemble de ces raisons, vous l'aurez compris, si le Gouvernement partage votre diagnostic et vos ambitions de régulation des géants de l'internet, il reste pour le moins réservé sur les modalités de mise en oeuvre figurant dans cette proposition de loi.

que technique dans ses détails et potentiellement complexe dans sa mise en oeuvre. Ce n'est pas sans rappeler nos débats de 2018 lors de la transposition de la directive sur le secret des affaires, en particulier sur la nécessité de concilier protection des intérêts économiques et liberté d'expression et d'information. L'actualité ne cesse de le démontrer pour le meilleur et parfois le pire, les technologies de l'information et de la communication, surtout lorsqu'elles sont mal maîtrisées- nous en avons eu récemment un exemple-, ne cessent de poser un défi à notre société, à nos pratiques quotidiennes, à nos rapports sociaux, à l'éducation de nos enfants et même à nos institutions. Le développement des appareils connectés- téléphones intelligents, tablettes, etc. -et des applications liées a innervé l'ensemble de notre économie au travers d'une offre impressionnante de logiciels, fournissant des services aussi variés que l'information journalistique, la banque, le paiement en ligne, des informations en temps réel sur le trafic et les transports en commun, ou encore les forums de discussion et l'organisation d'événements les plus divers. Ce développement a fait émerger de nouvelles possibilités et de nouveaux modes de consommation qui sont, au premier abord, plus faciles et surtout plus instantanés. Ils sont désormais bien ancrés dans le mode de vie d'une part croissante de la population, et les crises récentes- gilets jaunes, grève des transports -ont accentué cette tendance. Je n'en oublie pas pour autant nos compatriotes toujours exclus de l'accès à ces services, faute de bénéficier d'une couverture numérique dans leur territoire, ou simplement de savoir maîtriser l'outil informatique. À côté des bénéfices annoncés ou constatés pour les consommateurs, cette transformation s'accompagne d'une forte concentration de l'offre dans les mains de quelques entreprises très puissantes : les géants du numérique, principalement américains, qui tendent à acquérir une situation de monopole ou d'oligopole à cause des « effets de réseau » désormais bien connus. La croissance à deux chiffres du commerce en ligne depuis une décennie est une évolution majeure, et peut-être irréversible, qui entraîne des changements profonds dans la façon de consommer, bien sûr, mais aussi dans le monde du travail : progression spectaculaire du travail non salarié, et parfois remise en cause de droits attachés aux travailleurs. aux travailleurs. Je rappellerai également les enjeux du télétravail dans l'organisation du travail, un sujet sur lequel mon groupe a déjà fait des propositions. Face à cette tendance de fond, le principe de la liberté du commerce est paradoxalement remis en question. Plus grave, notre droit de la consommation et de la concurrence ne semble plus à même de répondre aux nouveaux enjeux. Les auteurs de la proposition de loi ont ainsi identifié des limitations dans le choix des applications permettant d'accéder au commerce en ligne, dans la capacité à passer d'un réseau social à un autre, ainsi que des limitations qui résultent des acquisitions prédatrices d'entreprises ou d'applications, pourtant innovantes, par des acteurs déjà installés- une logique classique, finalement, de la concurrence dans un contexte d'économie de marché avec effets de réseau. L'ambition du texte n'est donc pas mince ! Elle est de répondre à ces multiples défis, afin de redonner du pouvoir aux consommateurs à l'ère du numérique.

leur donnant davantage de compétences, conjointement avec le secrétariat d'État chargé du numérique. Des sanctions administratives sont prévues en cas de non-respect de leurs obligations par les fournisseurs, pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial. Par ailleurs, ces dispositions devront faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, en vertu d'une directive de 2015 sur la réglementation des technologies de l'information. Je salue également l'adoption, en commission, d'un amendement visant à instaurer la consultation de droit de la préalablement à l'établissement de nouvelles obligations en la matière. C'est une mesure protectrice des libertés. J'aurai donc peu de choses à ajouter sur un texte, rappelons-le, fort technique.

s'agissant de questions très complexes. C'est, me semble-t-il, un élément clé du succès d'un tel dispositif, dans la mesure où les utilisateurs non professionnels sont les premiers concernés. Monsieur le secrétaire d'État, j'attire particulièrement votre attention sur ce point

qui sont aussi des citoyens, sachent à quoi ils peuvent prétendre et comment ils sont protégés dans le cadre de leurs relations avec les plateformes. N'oublions pas que le modèle économique du numérique repose aussi sur la confiance. Cela étant, le RDSE votera en faveur de cette proposition de loi.

grâce au développement du numérique, le monde dans lequel nous vivons est en pleine mutation. Il est aujourd'hui à portée de clic, ce qui est à la fois une chance pour les consommateurs, mais aussi une source d'inquiétudes auxquelles il nous faut répondre pour protéger pleinement nos concitoyens. C'est une chance, puisque l'apparition de plateformes numériques et le développement des terminaux numériques intelligents que sont, aujourd'hui, les téléphones et, demain, l'ensemble des objets connectés créent des solutions innovantes pour les consommateurs et des opportunités nouvelles, notamment sur les plateformes d'achat. Les chiffres nous démontrent l'appétence des citoyens pour le cyberespace : le commerce en ligne a connu une hausse de 72 % entre 2014 et 2017, atteignant plus 2 300 milliards de dollars. Depuis sa création en 2004, Facebook est devenu le leader des réseaux sociaux. Il a d'ailleurs franchi un nouveau palier en 2017, avec 2 milliards d'utilisateurs actifs. Mais c'est aussi une source d'inquiétudes, car, face à la toute-puissance des géants du numérique que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, le risque de voir le consommateur entravé dans sa liberté de choix s'accroît au fur et à mesure que l'offre en ligne se développe. Il appartient donc au législateur de mieux protéger les consommateurs en garantissant leur liberté de choix sur les terminaux et en protégeant la libre concurrence des acteurs économiques sur le marché. Nous devons en effet permettre au consommateur d'installer les applications de son choix sur son smartphone et de changer de réseau social tout en gardant ses contacts. Nous devons également mettre fin à un certain nombre de pratiques qui limitent le libre choix du consommateur, comme l'impossibilité de désinstaller certaines applications préinstallées sur son smartphone. C'est dans ce contexte que nous examinons cette proposition de loi, adoptée à l'unanimité de la commission des affaires économiques. Nous partageons la volonté de renforcer les pouvoirs du régulateur national face à la toute-puissance des géants du numérique et l'objectif de ce texte, qui vise à rendre le pouvoir au consommateur en ligne. Je tiens à saluer le travail des rapporteurs, qui a permis d'enrichir le texte qui nous est présenté en suivant notamment les recommandations du Conseil d'État. Partant du constat, partagé, qu'il existe de nombreuses pratiques qui portent atteinte au libre choix du consommateur sur les smartphones, les trois mesures proposées permettront des avancées concrètes en la matière. Tout d'abord, il s'agit d'introduire une régulation sectorielle en vue d'assurer la liberté de choix du consommateur sur les terminaux. Ensuite, pour garantir la mobilité du consommateur sur les plateformes, le texte pose le principe d'interopérabilité des réseaux sociaux, afin de faciliter le passage d'un réseau social à un autre avec la possibilité d'interagir avec ses contacts tout en ayant changé de réseau social. Enfin, la lutte contre les concentrations prédatrices des Gafam est une priorité, afin de laisser l'innovation se développer, dans une logique de concurrence loyale des acteurs qui bénéficiera aussi aux consommateurs. L'Arcep, autorité de régulation en matière de télécoms, occupera un rôle central dans ce dispositif, en s'assurant que les pratiques mises en oeuvre sur les terminaux en vue de restreindre le choix des consommateurs ne sont pas injustifiées. Elle sera également dotée de pouvoirs de recueil et de traitement de l'information, d'un pouvoir de règlement des différends et d'un pouvoir de sanction des règles visant à protéger la liberté de choix des utilisateurs. La nécessaire régulation des géants du numérique ne date pas d'hier. De nombreux rapports ont en effet mis en lumière la nécessité de mettre en place une nouvelle forme de régulation de ces acteurs et l'État a pleinement conscience des enjeux actuels. C'est pourquoi, à la fin de l'année 2018, le Président de la République avait annoncé l'instauration d'une taxe sur les GAFA. Cette mesure, définitivement adoptée par le Parlement le 11 juillet dernier, a fait de la France le premier État à introduire en Europe une taxation de ce type, dans l'attente d'un accord à l'échelon international.

Il n'en demeure pas moins que les mesures prévues dans cette proposition de loi cosignée- je le rappelle -par l'ensemble des commissaires constituent des avancées réelles en faveur du libre choix des consommateurs dans le cyberespace. Ce texte démontre également la volonté du Sénat de travailler ensemble, de manière transpartisane, dans l'intérêt de nos concitoyens. Nous nous en félicitons et nous soutiendrons cette proposition de loi, tout en rappelant l'importance de parvenir rapidement à un accord au plan européen pour en garantir l'efficacité. La parole

La transformation d'internet en un vaste supermarché mondial pose la question de la liberté du commerce et de l'industrie en faveur de l'internaute, trop souvent transformé en simple consommateur du cyberespace. Les Gafam sont les grands bénéficiaires de cette croissance exponentielle du numérique commercial : s'est ainsi constitué un véritable oligopole de géants aux pouvoirs considérables sur nos vies, sur la maîtrise de nos destins individuels et collectifs. ont pu développer cette hyperpuissance par des stratégies variées, en particulier en bridant le libre choix de l'internaute par différents mécanismes, qui ne permettent pas une neutralité du Net.

Trois points sont en effet importants dans ce texte : assurer le libre choix sur les terminaux, garantir l'interopérabilité des plateformes, lutter contre les acquisitions prédatrices. S'agissant de la question des terminaux- nos smartphones et autres outils -, le Conseil national du numérique dès 2013 sur l'importance d'élargir la neutralité du Net à ces équipements : « Internet n'est pas seulement un réseau physique mais aussi [ ...] un ensemble de services. Il est inutile d'imposer la neutralité en amont si on ne change pas les règles en aval. » d'il y a sept ans ... Pendant ce temps-là, les géants du Net ont engrangé d'énormes profits et accru considérablement leur influence, en particulier en développant le web en silo.

Mais l'expérience de la taxation nous a montré que si quelques pays ne mènent pas l'offensive, avec des propositions déjà opérationnelles sur leur territoire pouvant être reprises par les autres, nous n'aurons que des heures et des heures de palabres

La question se pose aujourd'hui, avec la multiplication de règles du jeu de plus en plus détestables. Je prendrai les exemples de la loi du lynchage sur les réseaux sociaux, dont nous venons d'avoir, une fois de plus, des exemples révoltants avec les affaires Mila et Pavlenski la loi de la prétendue démocratie directe numérique, qui apparaît chaque jour un peu plus comme la tentative de meurtre de la démocratie représentative ; de la loi des rendements décroissants que je vous propose, selon laquelle la vitesse de fabrique du crétin digital augmenterait en proportion du temps passé sur les écrans et, enfin, de celle que nous allons combattre aujourd'hui sur l'initiative de Sophie Primas, la loi du plus fort. « Nous accomplissons des actes dont nous devenons les esclaves », disait Goethe au XIX siècle. Pourtant, à la fin du XX siècle, même les plus clairvoyants étaient peu nombreux à prédire que le bouleversement numérique mondial consacrerait l'émergence de nouveaux tyrans tout-puissants et qu'il le ferait insidieusement, car comme le dit le proverbe, « les bottes du diable ne grincent pas ». L'un des grands pionniers de l'internet, Robert Metcalfe, avait établi la loi qui porte son nom : l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Cette loi de l'effet réseau explique pourquoi les nouvelles technologies sont aujourd'hui régies par une poignée d'entreprises qui n'ont plus de concurrence sérieuse et peuvent imposer leurs lois contre les lois du marché et celles des États. C'est la tendance naturelle des réseaux d'absorber, comme un trou noir, tout ce qui gravite à leur périphérie et de réduire l'univers des possibles promis par internet à leur seul appétit monopolistique. Les Gafam n'ont au départ de puissance que celle que les citoyens leur donnent. Mais dès lors que leur place dans l'économie devient cardinale, les consommateurs et les entreprises n'ont plus d'autre choix que de se soumettre aux conditions léonines qu'ils imposent.

Il faut aujourd'hui non pas renverser nos valeurs et abandonner le libéralisme, mais adapter celui-ci à notre temps. Friedrich Hayek, qu'on critique plus qu'on ne le lit, écrivait Dans la conduite de nos affaires nous devons faire le plus grand usage possible des forces sociales spontanées, et recourir le moins possible à la coercition. [ ...] Il y a [ ...] une immense différence entre créer délibérément un système où la concurrence jouera le rôle le plus bienfaisant possible, et accepter passivement les institutions telles qu'elles sont. Rien n'a sans doute tant nui à la cause libérale que l'insistance butée de certains libéraux sur certains principes massifs, comme avant tout la règle du laisser-faire. » C'est pourquoi je tiens à saluer, au nom du groupe Les Indépendants, cette proposition de loi présentée par notre collègue Sophie Primas. Elle constitue l'aboutissement concret des travaux menés par la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, pilotée par mon collègue et ami Gérard Longuet. Je partage largement le constat de mes collègues : le meilleur moyen d'empêcher une casserole de déborder, c'est de la surveiller. Bien sûr, le choix de confier le sujet à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut paraître quelque peu virtuel devant l'ampleur de la tâche et du défi. Avec ses 170 agents et ses 27 millions d'euros de budget, ce serait pécher par excès d'optimisme que d'imaginer que l'Arcep aura les moyens de briser les monopoles d'entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse le PIB de nombreux pays. Mais ce serait baisser les bras que de ne pas confier au régulateur des moyens plus importants pour agir. La régulation en complément de la régulation, la détermination d'un principe d'interopérabilité des plateformes et la lutte contre les acquisitions prédatrices apparaissent à cet égard comme des pistes d'action indispensables pour engager un nouveau bras de fer avec les géants du numérique, après la taxe Gafam adoptée par le Parlement l'an dernier. Comme bon nombre d'entre nous, j'aimerais croire que nous sommes sur le point de voter ce qui pourrait être un du XXI siècle à la française. Mais à la différence des fameuses lois antitrust adoptées aux États-Unis à la fin du XIX siècle, les dispositions que nous allons voter ne concernent pas, pour l'essentiel, des entreprises implantées sur le territoire national. Il s'agit non plus de démanteler un réseau de chemins de fer à l'échelle d'un pays, mais de briser l'emprise de réseaux de données à l'échelle de la planète. Comme le font remarquer les auteurs de la proposition de loi, il s'agit donc de « cranter » aujourd'hui un sujet au niveau national pour le porter demain au plan européen. Car nous aurons besoin de nos partenaires européens pour mener à bien cette bataille. J'entends vos remarques, monsieur le secrétaire d'État, sur ce point, mais je vous répondrai qu'il est illogique pour le Gouvernement d'appliquer cette méthode en deux temps pour la taxe Gafam et de la refuser pour l'actuelle proposition de loi. Ce texte montre que notre assemblée est force de proposition pour s'attaquer aux grands défis de demain. Cela ne sera pas suffisant, mais il s'agit d'une étape importante. Nous avons combattu les dérives de l'internet hier par la fiscalité, nous les combattons aujourd'hui par la régulation et nous les combattrons- je l'espère -demain par la patrimonialité des données

De l'accaparation des données au verrouillage du système, certains géants du numérique s'affranchissent sans vergogne des règles des États, comme nous l'ont montré les affaires Snowden en 2013 ou Cambridge Analytica Dès 2013, le Sénat avait lancé l'alerte. En 2015, la rapporteure de la mission d'information relative à l'Europe au secours de l'internet, ma collègue Catherine Morin-Desailly, soulignait déjà combien la gouvernance de l'internet était un terrain d'affrontement mondial sur lequel se jouait l'avenir des valeurs européennes.

de la régulation économique dans le cyberespace. Elle vise à redonner du pouvoir au consommateur-internaute en définissant une régulation économique plus pragmatique et surtout plus réactive face aux pratiques évolutives des géants du numérique. Le déploiement de plateformes maîtrisées par un oligopole de géants du numérique a considérablement transformé les problématiques liées à l'exercice de la liberté du consommateur. En dépit des dispositions prises ces dernières années sur le plan du droit de la concurrence et de la consommation, le consommateur est devenu l'objet de quelques grands acteurs dominants qui cadrent les possibilités offertes, limitant la liberté de choisir les applications à installer sur son téléphone portable, ou encore la capacité à passer d'un réseau social à un autre. Cette liberté de choix est d'autant plus menacée que ces mêmes géants annihilent toute concurrence par des acquisitions prédatrices, qui éliminent ou neutralisent toute concurrence avant qu'elle ne leur fasse trop d'ombre, affectant de fait le libre choix du consommateur, mais aussi le potentiel d'innovation du secteur. L'économie numérique repose largement sur ce modèle de plateforme, de marché dit « biface », où le service facilite les interactions entre deux ensembles d'utilisateurs distincts, mais interdépendants

C'est l'effet de réseau, qui constitue la matrice de l'internet. Ce réseau se démultiplie sans connaître de frontières. Les plateformes ont accès à un marché mondial, recueillent des données en masse, et bénéficient d'économies d'échelle et de gamme sans précédent. Ces caractéristiques nouvelles et particulières favorisent la constitution d'une économie de la concentration et d'oligopoles. Ainsi, dès 2018, un tiers de l'humanité était sur Facebook et recourait à Android, le système d'exploitation de Google, et un cinquième utilisait celui d'Apple. Jusqu'à présent, le droit de la concurrence, qui réprime les abus de position dominante, les ententes, et assure le contrôle des concentrations, a pu dans une certaine mesure permettre aux autorités françaises et européennes de se saisir des enjeux relatifs au numérique.

Sept ans pendant lesquels les concurrents ont été éliminés, l'innovation bridée, les choix du consommateur encadrés. De son côté, la DGCCRF utilise le droit des pratiques restrictives de concurrence pour encadrer les relations commerciales des géants du Sur la base du constat, elle inflige des amendes. Elle s'assure de l'application des dispositions introduites dans le code de la consommation par la loi pour une République numérique de 2016. Mais toutes ces initiatives, qui sont autant d'aiguillons adressés à l'Union européenne pour renforcer le droit européen, c'est-à-dire qu'elles reposent sur des sanctions qui ne sont plus adaptées aux cycles d'innovation de plus en plus rapides et à la dynamique propre à l'économie du numérique. Il faut donc à présent confier à un régulateur les outils juridiques permettant de réagir rapidement aux pratiques des plateformes structurantes, avant

la régulation sectorielle, le principe d'interopérabilité des plateformes et la modernisation du droit de la concurrence. Je tiens à souligner les précautions qui ont été prises par le Sénat, notamment par son président, qui a saisi le Conseil d'État, afin de recueillir son avis sur cette proposition de loi et de s'assurer de sa portée portée juridique. Les remarques qui ont été formulées ont largement inspiré les rapporteurs dans les modifications qui ont été apportées en commission. Le groupe UC votera donc en faveur de cette proposition de loi, qui participe d'une stratégie globale de l'internet préconisée de longue date par le Sénat,

qui s'imposeront aux géants du numérique et permettront de contrecarrer la domination économique que certains cherchent à instaurer au détriment de la souveraineté des États. C'est en effet là, à mes yeux, que le bât blesse, monsieur le secrétaire d'État, et c'est peut-être la raison pour laquelle les États sont plus prompts à réagir que l'Europe. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en 2019, 49 millions de Français ont acheté des biens de consommation sur internet.

C'est dans ce contexte marqué par l'explosion du marché du e-commerce que l'État se révèle bien souvent démuni et impuissant pour élaborer et faire respecter une réglementation difficile à appliquer à des multinationales en position de monopole de fait.

parlait déjà de l'inquiétante extase que suscitait ce nouveau mode de communication et d'un espace public devenu un vide-ordures planétaire. Pour revenir à la taxation des géants du numérique, nous pourrions également égrener la litanie des tentatives infructueuses de légiférer sur ce sujet. La dernière taxe sur les GAFA, dont le Gouvernement nous a parfois tympanisés, a d'ailleurs été abandonnée face au risque de déclencher une guerre commerciale avec les États-Unis. Il n'empêche que cette étrange mise en scène traduit au moins les enjeux liés à ce sujet. Le rapport sénatorial de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique nous a alertés sur la nécessité de doter la France et l'Union européenne de mesures fortes et protectrices. En effet, la prédominance de certains acteurs et les enjeux économiques liés au e-commerce font peser un risque majeur sur les consommateurs. Songeons par exemple que Google et Facebook concentrent à eux seuls près de 75 % du marché de la publicité digitale en France. L'objectif n'est pourtant pas de faire fi de l'opportunité économique offerte par le numérique au marché français. Il n'est pas non plus question d'en brider l'essor. Pour autant, il est impératif de mettre en place des dispositifs à même de pallier les lacunes qui existent actuellement en matière de protection du consommateur sur le cyberespace. Aussi, la proposition de loi de Sophie Primas prévoit d'imposer une neutralité sur l'accès aux différents contenus les terminaux mobiles et de permettre par conséquent aux utilisateurs d'installer l'application ou le contenu qu'ils souhaitent. Il paraît anormal que les consommateurs soient privés de certaines applications selon qu'ils possèdent ou non tel ou tel type de téléphones, sous des prétextes commerciaux évidents. Je pense, comme cela a été dénoncé à plusieurs reprises, à Apple, qui dernièrement a refusé à ses utilisateurs la possibilité de bénéficier de titres de transport dématérialisés sur mobile. Au-delà du consommateur, ce sont les différents acteurs du e-commerce qui sont affaiblis par ce monopole. En effet, en 2019, la Commission européenne a été saisie d'une plainte du site de musical Spotify, accusant Apple de discrimination à l'encontre de son application sur l'App Store au profit de son propre service de musical. En renforçant le rôle et les pouvoirs de l'Arcep, cette proposition de loi permet de renforcer notre capacité de contrôle sur ces géants du numérique, et ainsi de préserver les consommateurs de pratiques abusives. En dépit des rodomontades, la France n'a que trop tardé sur ce sujet. En Allemagne, le Gouvernement s'est engagé sur un projet de réforme visant à adapter sa législation à l'économie numérique. Il est bien évidemment primordial d'oeuvrer à l'échelon européen, afin qu'une réglementation soit votée et appliquée à ce niveau. Mais cela ne doit pas nous empêcher de commencer à légiférer en ce sens. Je tiens à saluer le travail de la commission, qui a enrichi ce texte d'un nouveau chapitre sur la sincérité des interfaces utilisateur des plateformes numériques, afin de protéger le consommateur des pratiques abusives visant à obtenir son consentement de façon déguisée. Nous avons donc l'espoir que cette proposition de loi, si elle est adoptée, permette à la France de rattraper son retard et d'adresser un signal significatif aux entreprises du numérique, qui sont en position de quasi-monopole. La parole

je veux tout d'abord féliciter les rapporteurs pour leur travail sur ce texte, dont je me réjouis qu'il ait été déposé par la commission des affaires économiques à la suite des travaux de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique. La proposition de loi que nous examinons répond à une impérieuse nécessité, celle de protéger nos concitoyens vis-à-vis d'acteurs qui maîtrisent leurs données. Face au monopole des Gafam dans le cyberespace mondial, nous sommes pour l'heure confrontés à une stérilisation de cet espace, jadis bâti sur l'utopie d'une liberté de naviguer et d'entreprendre, à une dépossession des citoyens de leurs données personnelles et, surtout, à un vide juridique qu'il convient de combler. L'Europe s'est emparée de ces questions, mais la France doit être combative et force de proposition, comme elle l'a été avec la loi pour une République numérique, et comme elle l'est encore aujourd'hui pour ce qui concerne la fiscalité numérique ou la lutte contre les contenus haineux sur internet. Ce texte vise trois objectifs. Il vise, en premier lieu, à assurer le libre choix du consommateur sur les terminaux par l'introduction d'une régulation sectorielle. C'est une avancée importante, car l'économie de la donnée est d'ores et déjà un enjeu politique. C'est un capital pour nos pour nos entreprises, et la somme d'un vécu pour nos concitoyens, auxquels il faut apporter une protection. Il est donc normal de prévoir des outils de régulation, notamment dans une logique de supervision, pour lutter contre l'ultra-monopole des GAFA, qui réduisent la liberté de choix des consommateurs et empêchent les nouveaux acteurs économiques de les concurrencer. En l'espèce, cette proposition de loi donne les moyens à l'autorité de régulation, l'Arcep, de faire respecter les dispositions prévues, des sanctions pécuniaires. en second lieu, à établir l'interopérabilité des plateformes, c'est-à-dire faciliter la mobilité des consommateurs d'une plateforme à une autre ou d'un système d'exploitation à un autre. Aujourd'hui, l'interopérabilité reste très limitée. Or, si elle était assurée, cela ouvrirait davantage le champ de la concurrence et stimulerait l'innovation. L'interopérabilité, c'est le pouvoir de librement quitter une plateforme, sans perdre ses liens sociaux, et de continuer à communiquer avec ses contacts. C'est pour ainsi dire une liberté fondamentale, que chacun doit posséder dans le cyberespace, et que le politique doit garantir. C'est également un enjeu crucial de la capacité des acteurs de toutes tailles à faire émerger des offres compétitives sur le marché. En dernier lieu, ce texte vise à lutter contre les acquisitions dites prédatrices, en renforçant notamment notamment les missions de l'Autorité de la concurrence pour limiter la consolidation d'entreprises qui rachètent peu à peu tout un écosystème. C'est, par exemple, ce que Facebook a opéré avec le rachat d'Instagram et de WhatsApp. En l'état actuel du droit, l'Autorité de la concurrence n'a pas pu examiner ces rachats, car les sociétés ciblées ne réalisaient, aussi incroyable que cela paraisse, qu'un chiffre d'affaires limité, en tout cas inférieur au seuil de déclaration obligatoire au titre du droit des concentrations. C'est précisément ce dispositif qui doit évoluer, à l'échelon tant national qu'européen. Mais là où le rapport de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique allait plus loin, en proposant d'introduire un nouveau seuil basé sur une disproportion manifeste entre la valeur de rachat et le chiffre d'affaires réalisé par la société cible, la présente proposition de loi privilégie une information minimale par les entreprises systémiques. ce choix peut paraître frileux, témoignant de la volonté de rassurer les acteurs du numérique et de la crainte de les brider dans leurs initiatives. En réalité, cette solution, soutenue par ailleurs par l'Autorité de la concurrence, évite à celle-ci d'être saisie de nombreuses opérations sans incidence sur le marché et, réciproquement, aux entreprises concernées devoir déclarer une opération anodine. C'est une mesure de simplification assez souple, qui oblige néanmoins les entreprises systémiques à se mettre en relation avec le régulateur, ce qui est,, notre objectif. Enfin, les rapporteurs ont complété le texte avec des dispositions permettant de lutter contre les interfaces trompeuses, qui sont des pratiques déloyales, voire agressives, à l'encontre des consommateurs. Le groupe socialiste proposera de renforcer les moyens des régulateurs par des amendements concernant concernant l'auditabilité des algorithmes. Nous proposerons également de mieux définir la notion d'interopérabilité, ou encore les obligations de loyauté des fournisseurs de systèmes d'exploitation. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si certains jugent encore que ce texte n'est pas pertinent ou urgent, ou qu'il convient de laisser l'initiative d'un tel travail à l'Union européenne, je veux simplement rappeler un ordre de grandeur la capitalisation boursière des Gafam représente plus de deux fois celle du CAC 40 et dépasse les 4 000 milliards de dollars. Leur chiffre d'affaires est comparable à la totalité des recettes fiscales de notre pays. Autant dire que ces entreprises systémiques possèdent la puissance économique d'un État Il n'est plus temps de laisser un sujet d'une telle gravité s'enliser dans des questions de procédure juridique ou de tutelle. Sa complexité ne doit pas non plus nous arrêter. C'est à nous, hommes et femmes politiques, de doter l'État de moyens propres à freiner cet expansionnisme délétère et de protéger les intérêts et les droits de nos concitoyens, tout en favorisant l'innovation et la concurrence, non seulement nécessaires, mais saines pour tout marché. Il nous revient de défendre un modèle de société dans lequel l'être humain ne se résume pas à une somme de données à exploiter ni à des tendances à influencer. À ce titre, je me félicite de la saisine du Conseil d'État, qui a permis d'améliorer ce texte,

Cela ne fait qu'attester de leur position dominante, voire monopolistique. Ces dernières années, ces grands opérateurs ont mis en place le schéma suivant : ils rachètent des petites entreprises à fort potentiel, ce qui empêche l'émergence d'acteurs concurrents. Il est impossible de nier une concentration excessive du marché entre leurs mains, ce qui ne peut avoir qu'une incidence négative sur l'économie et la liberté de choix du consommateur, qui se voit enfermé dans un écosystème duquel il lui est quasiment impossible de sortir en raison des stratégies de ces grandes entreprises. C'est pourquoi ce texte ambitieux entend lutter contre ce phénomène, en renforçant les législations existantes, qui sont lacunaires. Une législation européenne dans ce domaine serait bénéfique, mais ce qui a été adopté à l'échelon de l'Union est timide. Or le milieu du numérique se caractérise par des cycles d'innovation très courts, ce qui permet de verrouiller le marché. Attendre une action de l'Union européenne ne fera donc que renforcer la position dominante de ces entreprises. Aussi, il est souhaitable que la France adopte d'abord une législation nationale, qui pourra ensuite servir de catalyseur au plan européen. Dans cette optique, cette proposition de loi introduit plusieurs nouveautés. Son but premier est de garantir le libre choix du consommateur. Pour ce faire, elle crée un droit d'accès et de diffusion aux informations et aux contenus, ainsi qu'un droit de fournir des applications et des services. Elle impose des obligations préventives aux entreprises, afin d'assurer ces droits. Elle interdit notamment de traiter des contenus de façon différenciée si cela est injustifié, de faire en sorte que des applications se trouvant dans la configuration initiale empêchent le consommateur de choisir des applications similaires provenant d'un autre fournisseur. également d'empêcher de façon injustifiée de supprimer des applications qui se trouvent dans la configuration initiale. Des dérogations sont prévues lorsque les entreprises sont confrontées à des obligations légales ou réglementaires, ou pour assurer la sécurité et le fonctionnement du terminal. Toutefois, et c'est tout à fait louable, la commission a décidé d'autoriser ces dérogations uniquement dans les cas où elles seraient strictement nécessaires aux entreprises. Cela permettra de limiter les abus. Le pouvoir de protéger les droits sera attribué à l'Arcep, qui pourra fixer des lignes directrices et édicter des recommandations sur le sujet. Elle aura aussi le pouvoir de recueillir des informations, un pouvoir de règlement des différends, ainsi qu'un pouvoir de sanction. Ce texte a également pour objet de permettre au consommateur de conserver ses contacts et liens sociaux sur d'autres plateformes que celles où ils ont été créés, en donnant à l'Arcep le pouvoir d'imposer des obligations tendant à rendre interopérables les services de communication en ligne lorsque cela lui paraît pertinent. À titre personnel, il me semblerait toutefois souhaitable de préciser sur quels critères se baser pour que cette mesure soit considérée comme pertinente. Des limites sont là aussi posées en cas de risque d'atteinte aux droits d'auteur, ainsi que dans le cadre de la protection des données personnelles. Enfin, les grandes entreprises seront obligées de prévenir l'Autorité de la concurrence de toute acquisition. Cette dernière aura la possibilité d'examiner des opérations qui seraient au-dessous des seuils de notification obligatoire si elle considère qu'elles sont susceptibles de faire peser un risque sur la dynamique concurrentielle. Des critères ont été déterminés, afin d'identifier les entreprises qui seront visées par cette obligation. De plus, et afin que l'Autorité de la concurrence soit à même de remplir sa mission, la commission a très justement décidé d'inverser la charge de la preuve en matière de contrôle des concentrations pour ces entreprises. Ce n'est plus l'Autorité de la concurrence qui devra démontrer que des règles ont été enfreintes, ce sont les entreprises qui devront prouver qu'elles ne sont pas dans l'illégalité.

c'est l'écosystème tel qu'il s'est construit. Nous sommes dans le modèle du capitalisme de surveillance, mes chers collègues. Très bien ! Nous sommes dans le modèle de l'attention, un modèle qui n'est pas durable ni soutenable.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 1 laisse la possibilité aux fournisseurs de systèmes d'exploitation de justifier d'éventuelles limitations au choix des consommateurs.

en le rendant plus restrictif, notamment en écartant la possibilité d'une restriction du choix des consommateurs pour le « bon fonctionnement de l'équipement terminal ».

le président, permettez-moi une petite déclaration liminaire, même si je ne réussirai probablement pas à convaincre la Haute Assemblée de suivre la position du Gouvernement. Vous l'aurez compris,

la commission. Le Conseil d'État a souligné que la possibilité de déroger aux obligations prévues par la proposition de loi pour des motifs de bon fonctionnement de l'équipement terminal était nécessaire pour préserver la faisabilité technique de la mesure. Supprimer cette exception conduirait à fragiliser la proportionnalité de ce dispositif.

Une récente affaire, dont ont été évoqués dans cette enceinte quelques tenants, a montré qu'à partir d'une information qui est faiblement repérable sur internet, Twitter et d'autres agissent comme des chambres d'écho pour lui donner une importance qui en fait, ensuite, quelque chose de tout à fait viral. Derrière cet effet chambre d'écho, il y a des algorithmes favorisant systématiquement l'information qui va, comme l'a dit très justement la présidente Morin-Desailly, faire fonctionner l'économie de l'attention. Plus une information peut attirer de l'attention, plus elle va être valorisée par les algorithmes.

car l'article 107 du code de la consommation prévoit déjà une obligation pour les plateformes d'informer les consommateurs sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels la plateforme permet d'accéder. C'est la raison pour laquelle nous vous en demandons le retrait, mon cher collègue.

Par exemple, le CSA s'est plaint à plusieurs reprises de ne pouvoir disposer des algorithmes que, pourtant, les opérateurs lui doivent. Vous ne pouvez pas me faire une réponse aussi lapidaire. Il faut que vous nous expliquiez, là, maintenant, quelle action systématique vous menez pour

quand le manquement en cause relève tout autant des atteintes à l'interopérabilité que des pratiques restrictives de concurrence, notamment l'avantage sans contrepartie ou le déséquilibre significatif,

à la pratique de ces plateformes au regard des critères d'interopérabilité figurant dans le texte, elle doit pouvoir se tourner vers le tribunal de commerce,

par le texte, qui permettra à tout utilisateur professionnel de saisir l'Arcep en cas d'atteinte à la neutralité des terminaux, et ensuite dans le cadre des nouveaux articles L. 109 et L. 113 du même code, grâce auxquels toute personne physique ou morale concernée pourra solliciter une sanction de la part de l'Arcep.

Je crois qu'il faut donner de vrais droits aux personnes morales ou physiques qui sont touchées, menacées, ou spoliées au regard des règles que nous sommes en train de mettre en place. Tout faire passer par l'Arcep réduit le champ

M. Alain Duran. Lorsqu'une personne fait une recherche sur internet ou sur un site de vente en ligne, les résultats de sa recherche subissent un référencement sur la base de critères propres à chaque site concerné. Ces critères ont une incidence directe sur le résultat des recherches que l'on effectue et, par conséquent, sur les produits que l'on achète. La question du référencement est donc centrale. La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé une obligation de loyauté : les plateformes doivent offrir une information claire sur les critères de référencement et indiquer les liens contractuels et capitalistiques qui peuvent exister avec les différents résultats référencés. mesure est d'éclairer le consommateur sur les raisons pour lesquelles certains résultats ont été mis en avant. Seules les plateformes en ligne sont concernées par cette obligation de loyauté, mais il nous a semblé que la question du référencement se pose également pour les terminaux mobiles, notamment les fameux « stores

à mettre en évidence les critères qui conditionnent le référencement des applications proposées et les liens capitalistiques qu'ils peuvent avoir avec les concepteurs de ces applications. Le sujet n'est pas anodin. À titre d'exemple, au premier trimestre 2018, les plateformes Google

La plupart de ces applications disposent d'achats intégrés. La question du libre choix est donc d'autant plus importante qu'elle implique une démarche d'achat. En conséquence, notre amendement vise à transposer l'obligation de loyauté applicable aux plateformes en ligne aux fournisseurs de système d'exploitation.

L'interopérabilité est une considération structurante pour la liberté des internautes ; la définition actuelle paraît donc insuffisante par rapport aux enjeux soulevés dans la présente proposition de loi.

conséquent parler d'interopérabilité d'un produit ou d'un système que lorsqu'on en connaît toutes les interfaces. Aussi, nous proposons de reprendre la définition de l'interopérabilité retenue dans le référentiel général d'interopérabilité. en effet le cadre de recommandations qui favorisent l'interopérabilité au sein des systèmes d'information de l'administration. Ces recommandations prennent en compte la nécessité de lever les barrières à l'interopérabilité, qu'elles soient d'ordre juridique ou technique. Nous proposons en conséquence, de définir l'interopérabilité comme la capacité que possède un produit ou un système dont les interfaces sont intégralement connues à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs, et ce sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre.

On nous oppose que la neutralité et l'interopérabilité du Net seraient déjà couvertes. Nous pensons que tel n'est pas le cas, puisque les opérations

d'une association agréée d'utilisateurs, ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner » les atteintes au libre choix et à l'interopérabilité des plateformes. Pour réparer collectivement le préjudice subi par les consommateurs devant les tribunaux, si la proposition de loi dont nous discutons devient loi, les atteintes à la neutralité des terminaux

d'un professionnel à ses obligations légales relevant ou non du code de la consommation « à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services » peut faire

Il se trouve que beaucoup de juristes qui travaillent sur ces sujets considèrent que la mise en oeuvre de l'interopérabilité et de la neutralité ne constitue pas une fourniture de services

autour du concept de « fourniture de services ». J'insiste sur ce point d'autant plus que les opérateurs que nous avons face à nous ne sont pas des enfants de choeur : ils vont déployer des batteries d'avocats pour tenter de trouver toutes les petites failles qui peuvent exister dans notre droit ! À l'étape où nous sommes, je pense donc qu'il est important de bien rappeler que les actions de groupe couvrent

Il est ainsi proposé de retenir une approche par indices, qui pourraient être mobilisés par l'Autorité de la concurrence pour caractériser l'importance de l'entreprise, sur les marchés français et européen. Cet amendement vise à clarifier et à préciser que l'Autorité de la concurrence devra recourir à un faisceau d'indices et non pas à un seul indice pour qualifier le caractère structurant d'une entreprise du numérique. de la commission ? Il s'agit d'une clarification bienvenue, car la qualification d'entreprise structurante doit provenir d'un faisceau d'indices ; un seul critère ne saurait être suffisant pour bien cibler les géants du numérique, les entreprises structurantes. La commission émet donc un avis favorable

Mme Viviane Artigalas. Les algorithmes prennent une importance considérable dans l'économie numérique et sont au coeur du fonctionnement de certaines entreprises. Leur transparence et leur fonctionnement font cependant débat et posent de nouvelles questions aux régulateurs. S'agissant des opérations de concentration et de pratiques anticoncurrentielles, il existe un risque que les algorithmes facilitent ou autorisent des comportements contraires au droit de la concurrence. Il faut désormais s'interroger sur les usages commerciaux des algorithmes, les algorithmes de prix, ou encore sur les risques de collusion horizontale. Il paraît essentiel d'aborder dans ce texte la question de l'auditabilité des algorithmes, comme le Sénat l'a fait récemment dans le cadre des débats sur la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Pour s'assurer que les algorithmes n'aient pas d'effets néfastes sur le fonctionnement concurrentiel des marchés, les autorités publiques compétentes, en l'espèce l'Autorité de la concurrence, doivent avoir une connaissance approfondie des systèmes algorithmiques utilisés par les plateformes numériques.

prévue répond d'ailleurs à l'une des recommandations de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique. J'ajoute que ce même dispositif a été proposé par voie d'amendement dans le cadre de la discussion de la

pour mutualiser ces compétences rares et chères que sont celles des, les spécialistes en intelligence artificielle, au bénéfice des administrations, mais également des autorités indépendantes. Ce de cette compétence et de la capacité technique et technologique à vérifier ce qui se passe au sein des entreprises du numérique, notamment des réseaux sociaux, à travers leurs algorithmes et les dispositifs qu'elles déploient. En l'espèce et juridiquement, l'alinéa 4 de l'article L. 450-3 du code de commerce autorise déjà les agents concernés à recueillir tout renseignement utile pour les besoins de l'enquête, sans qu'il soit nécessaire de préciser que tel est également le cas pour les données relatives aux algorithmes.

C'est bien de créer un service, mais il va falloir dégager des moyens financiers considérables. Nous constatons bien que tous les ingénieurs et mathématiciens français, qui sont particulièrement doués en matière d'algorithmes, sont recherchés par les Gafam

qui gouverneront nos choix. L'investissement dans les nouvelles technologies et la recherche, qui est encore largement insuffisante, devra être

les envies du consommateur par des recommandations personnalisées. On le voit tous les jours sur les réseaux sociaux. L'utilisation des algorithmes dans le secteur du e-commerce peut mener à des pratiques pouvant être considérées comme déloyales, voire trompeuses ou agressives, à l'encontre des consommateurs. Comme le souligne le rapport de la commission, il s'agit de pratiques auxquelles nous sommes tous confrontés au quotidien : des cases pré-cochées relatives au paiement d'une assurance que l'on ne souhaite pas, ou encore la désinscription à un service quasiment impossible à trouver. À ce titre, l'article 8 A, introduit en commission par les rapporteurs, est très intéressant et permet de lutter contre les interfaces trompeuses. Les grandes plateformes devront s'abstenir de proposer de telles interfaces, sous peine de sanction administrative prononcée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cet amendement vise donc à renforcer les moyens d'action de la DGCCRF,

en effet déjà les agents de la DGCCRF à avoir « accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. » Cette rédaction permet une adaptation à toute évolution technique ultérieure, alors qu'un excès de précision nous semble comporter le risque de limiter le champ d'application de l'article, d'autant que la rédaction proposée n'apporterait à notre sens rien de plus que ce qui est déjà possible aujourd'hui. Pour cette raison, le Gouvernement demande le retrait de cet

Il s'agit donc d'une question de principe et non de moyens. C'est pourquoi il est proposé d'étendre l'interdiction prévue par le présent article à l'ensemble des opérateurs et pas seulement aux grands opérateurs.

Les dispositions de l'article 8 A, que cet amendement vise à compléter, sont redondantes avec les dispositions déjà prévues par le code de la consommation pour les pratiques commerciales trompeuses. Cet article ne fait que répéter le droit en vigueur dans un cas particulier. Le comportement visé est en effet interdit de façon générale et peut être très lourdement sanctionné. Altérer l'autonomie de décision ou le consentement du consommateur par des artifices techniques est un agissement grave et une pratique commerciale trompeuse. Pour rappel, cette pratique est passible dans le droit actuel d'une amende potentiellement très élevée- elle peut être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel en fonction de l'avantage tiré du délit -et d'une peine d'emprisonnement de deux ans, selon les articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation. Pour rappel encore, l'interdiction et la sanction de ce type de pratique résultent de la directive européenne de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, qui est d'harmonisation maximale. Cette interdiction ne se limite pas aux grands acteurs, car ces pratiques déloyales ne sauraient être tolérées dans aucun cas.

2016 pour une République numérique, pour assurer la protection des consommateurs. Il s'agit en effet de donner aux utilisateurs d'internet une information claire sur les critères de référencement et d'indiquer les liens contractuels et capitalistiques qui peuvent exister entre les différents résultats référencés. Concrètement, l'objectif est d'éclairer le consommateur sur les raisons qui font que certains résultats de sa recherche ont été mis en avant. La loi pour une République numérique a posé les premières bases d'une régulation proactive des acteurs systémiques du numérique. numérique. « Dresser rapidement le bilan de l'application des principes de loyauté et de transparence des plateformes » fait partie des recommandations de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique présentées le 1 octobre cet amendement tend à reprendre cette recommandation en demandant au Gouvernement la présentation d'un rapport sur le respect et les conditions d'application de l'obligation de loyauté et de transparence.

adoptées dans le cadre de la loi pour une République numérique. Cet amendement s'inscrit donc dans ce cadre. Cela étant, la commission va en rester à la jurisprudence

visées. Compte tenu de l'information disponible, la demande me paraît satisfaite. En effet, dans le cadre de l'application de la loi pour une République numérique, la DGCCRF réalise des enquêtes nationales pour veiller à la bonne application de ces dispositions.

élevé. Seule une plateforme s'est rapidement mise en conformité avec la réglementation sur un total de 29 plateformes contrôlées, ce qui a donné lieu à 22 injonctions et à 4 avertissements.

Mme Primas et ses collègues de cette proposition de loi, qui arrive au bon moment,

Le scrutin est ouvert.